Monsieur le président,

La séance est reprise. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires sociales a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement.

Nous reprenons l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Vous me rétorquerez qu'il n'est pas besoin de surcharger la législation. Pourtant, dans le même temps, le Gouvernement a fait adopter une loi très médiatisée pour interdire le téléphone portable à l'école, une interdiction déjà inscrite dans le règlement intérieur de 90 % des établissements scolaires.

santé, compilant 350 études indépendantes, a reconnu en 2015 ce pesticide massivement utilisé comme un « cancérigène probable ». Le principe de précaution aurait déjà dû amener à l'interdire. Contrairement à ce que n'a pas manqué de nous opposer la majorité sénatoriale, c'est à nos agriculteurs, à leur santé que nous pensons en premier lieu, afin justement qu'ils puissent prendre leur retraite. Porter un masque à gaz pour pulvériser n'est pas anodin sortir de sa journée de travail avec des rougeurs et des maux de tête non plus. Mais ce n'est pas tout : l'impact du glyphosate est une catastrophe écologique. L'air, les sols et l'eau subissent une contamination généralisée. L'impact sur la biodiversité est certain. Les insectes, les oiseaux, les vers de terre, déjà menacés, sont un peu plus décimés par l'usage quotidien de ce produit. Cela entraîne un cercle vicieux. Les sols sont moins bien nourris cela nous force à utiliser de plus en plus de produits de synthèse pour faire pousser nos fruits et nos légumes, ce qui en retour abîme un peu plus nos sols. Qui pis est, à utiliser sans arrêt le glyphosate, nous favorisons la sélection des herbes et des insectes les plus résistants, plus dangereux pour nos cultures et plus difficiles à combattre, à l'aide de produits toujours plus nocifs. On ne s'en sortira certainement pas avec le recours à d'autres solutions chimiques, sans cesse invoqué comme un mantra. Une seule alternative existe : amorcer rapidement une transformation globale de notre modèle agricole. La

Cet amendement vise donc à interdire l'utilisation de ce produit à compter du 1 janvier 2021, avec de très rares dérogations jusqu'au 1 janvier 2022 pour les usages et les pratiques agricoles qui, sans ce produit, pourraient être en situation d'impasse au regard des leviers d'action et des connaissances actuels. Le glyphosate a été classé comme cancérogène probable sur le cancer, le CIRC, organe dépendant de l'OMS, en 2015. Depuis cette date, cette classification a fait l'objet de nombreuses controverses, voire de revirements, mais le doute sur sa toxicité demeure plus que jamais. agronomique, l'INRA, démontre que de nombreuses alternatives au glyphosate sont d'ores et déjà disponibles, notamment pour les grandes cultures, la viticulture et l'arboriculture, qui sont les filières les plus consommatrices de ces produits. En 2017, la France a voté contre le renouvellement pour cinq ans de l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate, en optant pour un délai plus court de trois ans. Nous n'avons malheureusement pas été entendus. Afin de sensibiliser les consommateurs à l'arrêt progressif de l'utilisation du glyphosate, cet amendement prévoit par ailleurs un étiquetage de l'ensemble des produits commercialisés en France, qu'ils soient bruts ou transformés, qui ont été traités par un produit contenant cette substance. Il s'agit non pas d'une utopie ou d'une lubie, mes chers collègues, mais bien de la concrétisation d'une promesse de campagne du Président de la République. Il s'agit désormais de passer de la parole aux actes.

rectifié. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, braque ou pas braque, je vous salue tous ! Nous souhaitons voir inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi.

Équilibre dans la temporalité, tout d'abord : elle est en accord avec la parole présidentielle et la prise de position de la France sur l'arrêt de l'utilisation du glyphosate en 2021, tout en prévoyant des mesures transitoires jusqu'en 2023. Cela va dans le sens

Équilibre dans la mesure, ensuite : le dispositif de l'amendement prend en compte les réalités économiques du secteur agricole et des filières en jeu, et il évite les effets néfastes d'une distorsion de concurrence.

d'exploitation des terres. C'est l'occasion pour notre pays d'être à la pointe de l'innovation dans ce secteur. Équilibre, enfin, dans une perspective de santé publique : s'il faudra sûrement remettre à plat la méthodologie

pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents de travail, l'INRS, rappelle que 30 % des maladies professionnelles reconnues en Europe seraient d'origine chimique. Telles sont les raisons

Le Président de la République a pris l'engagement de réussir cette sortie du glyphosate en trois ans au lieu de cinq, sans laisser les agriculteurs sans solution. Un groupe de suivi de cette sortie a été mis en place, le Gouvernement s'étant emparé de cette question. Le glyphosate a été classé comme cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS. L'Agence européenne de sécurité des aliments tout comme l'Agence européenne des produits chimiques ont pour leur part estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'exposition au glyphosate et le développement de cancers chez les humains. travail, déclare ne pas disposer de preuves suffisantes pour classer le glyphosate comme substance cancérigène. Néanmoins, dès qu'elle dispose d'éléments probants, elle agit, comme ce fut le cas lorsque l'effet cocktail entre le glyphosate et l'un de ses adjuvants, la tallowamine, s'est déclaré. Elle a alors retiré l'autorisation de mise sur le marché de tous les produits associant ces deux substances.

20 % des surfaces agricoles seraient consacrées à l'agriculture biologique en 2020. Aujourd'hui, nous en sommes à 6,5 %. Nous avons fixé un objectif ambitieux de 15 % à l'horizon de 2022, et il faudra le tenir.

l'agriculture de conservation et la culture des légumes pour l'industrie -, il n'existe pas d'alternative aujourd'hui. Mais personne ne sera laissé sans solution.

En effet, la stratégie du Gouvernement repose sur un engagement de tous : les agriculteurs, bien sûr, mais aussi l'aval des filières. Nous ne souhaitons pas faire peser tout le poids de cette responsabilité sur les agriculteurs. Nous voulons au contraire permettre une transition durable et mature, en impliquant à la fois les industriels et la distribution, que nous avons réunis, avec Nicolas Hulot, il y a huit jours. Nous avons demandé à chacun des acteurs de nous faire part, sous trois semaines, de leurs engagements en matière de réduction des usages du glyphosate et de valorisation des produits sans glyphosate.

l'ACTA. Le Gouvernement a fait le choix d'en appeler à la responsabilité de tous les acteurs, qui ont exprimé leur totale adhésion à cette démarche. Pour cette raison, je suis défavorable aux amendements qui ont été présentés. L'inscription dans la loi ferait peser sur les seuls agriculteurs les surcoûts liés à la diminution de l'utilisation du glyphosate. Or chaque maillon de la chaîne- producteur, distributeur, transformateur -doit contribuer à cet effort. Elle affaiblirait en outre la dynamique dynamique recherchée par le Gouvernement, qui est fondée sur la mobilisation, la responsabilisation de tous les acteurs, la confiance, le pragmatisme, la ténacité, une volonté sans faille. Vous serez bien évidemment tenus informés

Étude après étude, ces dangers se révèlent plus évidents. En 2002, des chercheurs de la station biologique de Roscoff établissent le caractère cancérigène probable du glyphosate sur l'embryon d'oursin. En 2012, un bond du nombre de tumeurs et de la mortalité chez les rats exposés au Roundup est observé par le Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique. En 2015, enfin, c'est au tour du Centre international de recherche sur le cancer, rattaché à l'OMS, de définir le glyphosate comme un cancérogène probable pour l'homme. Dans les pays où le glyphosate a été utilisé le plus intensivement, sa toxicité fait peu de doute. En Argentine, où l'agriculture intensive est tout particulièrement pratiquée, son introduction s'est accompagnée d'une explosion du nombre de cancers et de malformations. Le Sri Lanka, il y a quelques années, a interdit le glyphosate, car il causait des maladies rénales chroniques pouvant être fatales, surtout avec un effet cocktail avec les métaux lourds. Nous reconnaissons les difficultés d'une interdiction du glyphosate pour les agriculteurs dont le mode d'exploitation est lié à l'emploi de ce pesticide, y compris en termes de matériels agricoles utilisés, mais les enjeux de santé sont tels qu'il faut changer. Cette dépendance a, de toute façon, de graves inconvénients. Elle a des effets délétères, notamment sur le sol : ravinée par les pluies, la couche fertile s'en va, ce qui provoque des coulées de boue, et la

L'exigence des Européens, c'est d'avoir aussi confiance dans les experts qui nous éclairent. Nos récents débats sur le glyphosate, les perturbateurs endocriniens montrent la nécessité d'évaluation scientifique européenne plus transparente, plus indépendante, d'une recherche mieux financée qui permet d'identifier les risques et de proposer des alternatives. C'est indispensable. Nous avons aujourd'hui des débats politiques qui, parfois, cherchent à se substituer au débat scientifique. C'est la science qui doit éclairer la dangerosité, mais qui doit ensuite, de manière indépendante, transparente, indiquer les alternatives possibles scientifiquement démontrées.

des paroles de sachants ou des paroles d'autorité ni ne doivent accepter de laisser la place à une parole publique qui est celle de lobbies, d'intérêts industriels et qui construisent l'opacité sur des décisions collectives qu'attendent nos concitoyens.

le débat, dans notre pays, tournait autour de la date et du délai jugés les plus judicieux pour l'interdiction du glyphosate. Aujourd'hui, nous en sommes finalement à déterminer si, oui ou non, il est scientifiquement prouvé que ce produit est néfaste pour la santé et s'il faut réellement songer à l'interdire

importants. Soyons raisonnables, dépassionnons un peu le débat, et nous verrons que, demain, les choses iront progressivement

Ainsi, la seule agence à déclarer le glyphosate comme probablement cancérigène est le CIRC. D'autres agences, telles que l'OMS, l'ECHA ou l'EFSA, ont pris la position inverse. Toutes se sont fondées sur des compilations d'études.

quatre-vingt-seize scientifiques indépendants reprochent à l'EFSA de prendre en compte des études financées par des industriels, dont seuls les résultats sont accessibles. Or, si l'on ne connaît pas la méthodologie d'une étude, il est impossible de savoir si elle est solide, si elle comporte des biais, quels seuils de significativité ont été retenus.

l'alimentation n'est pas le seul facteur d'exposition, le cancer n'est pas la seule pathologie humaine et l'humain n'est même pas seul concerné, puisque la toxicité du glyphosate pour les animaux a été montrée par diverses études. Surtout, « peu probable » ne veut pas dire « certain

En l'état actuel des connaissances, nous ne disposons d'aucun élément qui pourrait permettre un retrait immédiat des AMM des formulations à base de glyphosate.

Le scrutin est ouvert.

Avant d'être autorisé, un produit phytosanitaire doit passer un certain nombre de tests réglementaires attestant de sa sûreté pour la santé et l'environnement. Dès lors, c'est l'intégrité des procédures d'évaluation du risque présenté certains pesticides pour les abeilles que nous souhaitons renforcer par cet amendement. En effet, ces protocoles ont été conçus par des groupes d'experts noyautés par l'industrie agrochimique. Deux ONG ont passé en revue douze méthodes ou pratiques standards utilisées par les agences d'expertise publiques pour évaluer les risques sanitaires ou environnementaux présentés par les produits phytosanitaires : dans 92 % des cas examinés, les techniques en question ont été codéveloppées par les industriels concernés, directement ou indirectement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2013 l'EFSA a produit, à la demande de la Commission européenne, des lignes directrices afin d'évaluer l'impact des pesticides sur les abeilles selon un protocole plus indépendant. Dans le même temps, l'OCDE a produit une série de nouveaux protocoles, validés internationalement, pour évaluer plus en détail l'impact des produits phytopharmaceutiques sur les insectes pollinisateurs. Toutefois, la France utilise encore des protocoles antérieurs, qui ne permettent pas d'évaluer l'impact effectif des pesticides. L'importance de la pollinisation, au coeur de la nature et de ses processus de reproduction, et le rôle joué par les abeilles et autres pollinisateurs pour l'équilibre des écosystèmes ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi il est important de suivre toute recommandation européenne ou internationale en la matière, en mettant notre législation en phase avec celle-ci. Nous souhaitons ainsi compléter l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits, en spécifiant que les dernières lignes directrices produites en matière de préservation de la biodiversité et des insectes pollinisateurs, au niveau européen et international, doivent être prises en compte et appliquées dans le cadre des procédures d'homologation

pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Depuis sa publication, il a fait l'objet de nombreux échanges entre les experts des États membres. Ces discussions n'ont pas encore abouti et le document n'a toujours pas été validé par l'ensemble des États membres au niveau européen.

L'objet de cet amendement est de formaliser l'obligation de prévoir l'inclusion, dans les formations nécessaires à l'obtention du certificat permettant l'utilisation, la vente ou le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques-

Ils peuvent souvent être préparés par des agriculteurs ou par de petites entreprises et appartiennent au domaine public. Ils permettent aussi, ce qui est important, l'autonomie des agriculteurs. sont efficaces et largement utilisés sur le terrain. Dans ces conditions, pourquoi ne pas prévoir de former à grande échelle les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques à

le recours aux antibiotiques vétérinaires. Toutefois, la directive européenne de 2001 précise que la publicité auprès du public, y compris les éleveurs, pour les médicaments vétérinaires délivrés sur prescription, ce qui est le cas des vaccins, est interdite. Les négociations en cours au niveau européen ont prospéré ; le projet de texte sur le médicament vétérinaire comporte bien une autorisation de la publicité pour ces vaccins auprès des éleveurs. Il faut s'en réjouir, mais le texte n'est pas encore formellement adopté et il ne pourra en outre entrer en application qu'après un certain délai.

de la Charte de l'environnement prévoit que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques De plus, une décision de la Cour européenne de justice du 23 novembre 2016 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement a précisé que la notion d'« émissions dans l'environnement », au sens de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, inclut notamment le rejet dans l'environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive précisant que les États membres ne peuvent prévoir qu'une demande d'accès à des informations relatives à des émissions dans l'environnement soit rejetée s'applique bien aux informations relatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait, les scientifiques et les citoyens n'ont pas accès aux données relatives à l'utilisation effective de ces produits qui sont détenues par l'administration. Le présent amendement prévoit d'appliquer à ces données la même transparence que celle qui a été instituée par la loi pour la République numérique pour de très nombreuses données publiques. Quel

L'idée est de préserver l'indépendance de l'activité de conseil, en particulier à l'égard des intérêts commerciaux d'une entreprise qui assurerait les deux activités

Le conseil est aujourd'hui majoritairement dispensé par les agents commerciaux des coopératives, qui sont intéressées à la fois à vendre davantage d'intrants- semences, engrais, pesticides -et à collecter un volume de récolte maximal.

il ne s'agit plus de passer notre temps à contester le fait que l'utilisation des produits phytosanitaires menace la santé des consommateurs et des agriculteurs, ainsi que la biodiversité, il s'agit de savoir comment nous nous mettons collectivement en situation de traiter ce problème. Nous soutenons pleinement la trajectoire ambitieuse du Gouvernement pour parvenir à une réduction efficiente de l'utilisation des produits phytosanitaires et nous voulons reprendre l'engagement du Président de la République sur la séparation capitalistique des activités de conseil et de vente. Certes, il apparaît aujourd'hui que les activités de vente et de conseil sont liées par nature. Cependant, cette situation crée nécessairement un conflit d'intérêts. Nous devons donc prendre nos responsabilités pour faire évoluer le paysage socioéconomique agricole. Cette séparation capitalistique permettra de mettre en place un conseil indépendant, moteur d'une stratégie efficiente permettant réellement l'amélioration des rendements, la protection des exploitations, voire la transition

Il est aujourd'hui nécessaire que les agriculteurs comprennent que le conseil n'est pas gratuit. C'est une réponse au défi sociétal d'une agriculture moins dépendante des produits phytosanitaires. Une nouvelle France agricole a été promue lors des États généraux de l'alimentation, puis au travers de ce projet de loi,

L'activité de conseil, séparée de l'activité de vente, doit s'inscrire dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Nos débats des derniers

travaux de la commission, les coopératives et le négoce agricoles vont continuer à assurer tout à la fois les activités de vente et celles de conseil spécifique. Celui qui détermine l'acte d'achat de pesticides par les agriculteurs

pour les produits phytopharmaceutiques. Je considère que c'est une étape nécessaire pour changer de modèle agricole. La personne qui vend, et qui a donc vocation à vendre toujours plus, ne peut pas être la même que celle qui apporte un conseil sur les produits, surtout à l'heure de l'agroécologie et de la nécessité de réduire l'usage des produits phytosanitaires.

Quand une maladie végétale se déclare, l'agriculteur doit, dans l'urgence, savoir vers qui se tourner, et c'est le plus souvent à son fournisseur de solutions, à savoir sa coopérative ou le négoce, qu'il s'adresse.

Enfin, la commission a précisé que, dans la perspective d'un conseil individuel réellement stratégique, celui-ci doit être pluriannuel, car l'agriculteur a besoin d'un appui sur plusieurs années pour favoriser la mise en oeuvre d'une stratégie de long terme et de lutte intégrée., intégrée., un conseil indépendant annuel entraînerait une charge excessive pour nos agriculteurs. La commission estime donc que la rédaction actuelle du texte est équilibrée et pragmatique, car elle assure un compromis entre la nécessaire évolution des activités de vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques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

est ainsi libellé : La parole est à M. le ministre. Il s'agit de rétablir la fixation par ordonnance de l'obligation, pour les opérateurs de la restauration collective, d'un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l'approvisionnement durable.

Aujourd'hui, ces variétés, issues de mutagénèse, et non de transgénèse, ne sont pas reconnues comme et sont donc exclues du champ d'application de l'interdiction des OGM. Ainsi, il est impossible de savoir combien d'hectares sont plantés en colzas et en tournesols génétiquement mutés pour tolérer des herbicides. Cependant, il semble bien que les surfaces progressent : le ministère de l'agriculture considère que 37 000 hectares de colza muté tolérant un herbicide ont été semés en 2016. du tournesol tolérant un herbicide occupait 160 000 hectares en 2016, selon Agrodistribution. Or ces variétés posent de nombreux problèmes, sans pour autant présenter d'avantages agronomiques.

peu de différences de rendement entre variétés tolérantes et non tolérantes. Décider un moratoire semble ainsi pleinement justifié, à la fois pour les agriculteurs, qui ne tirent pas de rendement supplémentaire de ces récoltes, et pour la santé publique, puisque le risque est accru pour la qualité de l'eau. Par ailleurs, cet amendement vise à répondre à une demande massive

? L'usage d'antibiotiques d'importance critique a été strictement encadré. Un décret de 2016 interdit aux vétérinaires de les utiliser en traitement préventif individuel ou collectif chez des animaux sains, même exposés à une maladie infectieuse. Les antibiotiques critiques listés peuvent, en revanche, être prescrits pour des traitements curatifs, c'est-à-dire chez des animaux malades, ou métaphylactiques, à savoir chez des animaux du même lot qui présentent une forte probabilité d'infection. Leur prescription par le vétérinaire est soumise à plusieurs exigences, notamment un taux élevé de morbidité, l'absence d'autres médicaments efficaces et une durée limitée de traitement. Ils sont donc utilisés en dernier recours, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution, et ne contribuent plus à l'antibiorésistance. Interdire ces traitements, c'est mettre en péril des exploitations dont l'élevage est confronté à une maladie qui ne peut être soignée par d'autres moyens. De plus, séparer la prescription de la vente d'antibiotiques pour les vétérinaires reviendrait à mettre en difficulté un certain nombre de vétérinaires ruraux qui, nous le savons,

prévoit que les missions des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté comportent obligatoirement un volet consacré à l'éducation alimentaire et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ces comités réunissent, sous la présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves. Actuellement, ils se voient confier quatre missions, en matière d'éducation à la citoyenneté, de prévention de la violence, d'aide aux personnes en difficulté et de programme d'éducation à la santé, à la sexualité et à la prévention des comportements à risques. Notre amendement tend à élargir le champ de ces missions en ajoutant un volet consacré à l'alimentation et le gaspillage alimentaire. Nous considérons en effet que les habitudes et comportements alimentaires s'ancrent dès le plus jeune âge. monsieur le rapporteur. Les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté ont été créés par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Ces comités sont institués au niveau académique, au niveau départemental et au niveau de l'établissement. Ils associent variablement des acteurs de la communauté éducative, aux fins de permettre la définition de parcours d'éducation à la santé et à la citoyenneté et de lutter contre les exclusions. Je partage la préoccupation de mes collègues : il ne serait pas inutile, dans le cadre d'un parcours de construction de la citoyenneté des élèves, que ces comités comprennent un volet relatif au gaspillage alimentaire. Néanmoins, cette formulation me gêne à plusieurs titres.

Par la suite, en novembre 2016, une résolution adoptée par le Sénat a conclu à la nécessité impérieuse d'acclimater les normes agricoles européennes au milieu tropical. En effet, ces normes trouvent leur origine, pour l'essentiel, dans des règlements européens, qui, à la différence des directives, ne nécessitent pas de transposition. Il s'agit donc, avec cet amendement, de parvenir à lister et à adapter les normes européennes qui auraient pu être acclimatées et qui ne l'ont pas été. Cela répond d'ailleurs au voeu du Président de la République, qui déclarait à Cayenne, le 27 octobre dernier, que « nous devons collectivement engager un travail sur l'adaptation des normes communautaires à ces territoires dont les contraintes et l'environnement sont spécifiques ». C'est d'ailleurs le même travail que nous allons mener concernant les normes nationales, qu'elles soient constitutionnelles ou législatives, dans le cadre des assises des outre-mer.

trouvent leur origine pour l'essentiel dans des règlements européens, malgré le maintien de compétences nationales importantes dévolues à l'ANSES et au ministre de l`agriculture ». Par la suite, en novembre 2016, une résolution du Sénat de M. Magras,

Les normes applicables à l'agriculture des régions ultrapériphériques françaises en matière sanitaire et phytosanitaire trouvent leurs origines, pour l'essentiel, dans des règlements européens, qui ne sont vraiment pas adaptés

présenter l'amendement n° 119 rectifié. Cet amendement vise à préciser la définition légale de l'agroécologie, dans le cadre de la parution d'un décret du Conseil d'État. Selon la définition retenue par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, l'agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie, tout en visant à diminuer les pressions sur l'environnement et à préserver les ressources naturelles. Il s'agit d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production, en maintenant ses capacités de renouvellement. L'agroécologie implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l'exploitation agricole dans son ensemble. C'est grâce à cette approche systémique que les que les résultats techniques et économiques peuvent être maintenus ou progresser, tout en améliorant les performances environnementales. L'agroécologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée. Le rôle de la biodiversité comme facteur de production en sort renforcé, voire restauré. L'agronomie est au centre des systèmes de production agroécologique. De solides connaissances dans ce domaine sont indispensables, tant pour les agriculteurs que pour leurs conseillers. La dynamique des eaux, les cycles biogéochimiques, les épidémies ou les pullulations de ravageurs sont liés à des échelles plus vastes que celles des parcelles cultivées. Aussi le passage à l'agroécologie doit-il également être pensé à l'échelle des territoires.

l'amendement n° 216 rectifié. Si l'agroécologie fournit un nouveau cadre de développement pour l'agriculture française, qui ambitionne de passer d'une logique d'exploitation du sol et des autres ressources naturelles à une logique de gestion d'écosystèmes cultivés, elle reste aussi un concept sans définition unique et sans reconnaissance officielle, en particulier au niveau européen. Il existe ainsi un risque important qu'une dénomination sans aucune valeur juridique permette à l'agriculture conventionnelle de valoriser une modification minimaliste de ses pratiques, tout en entretenant le flou quant à sa proximité avec l'agriculture biologique, qui correspond, elle, à des exigences élevées, définies par un règlement. Dans ces conditions, afin que l'agroécologie recouvre un réel changement des pratiques agricoles, cet amendement vise à ce que soit élaboré un cahier des charges précis et ambitieux en termes de croissance de la biodiversité, d'amélioration de la qualité des sols, d'économie d'eau pour l'irrigation, de reconstitution de paysages ruraux de qualité, de réduction des intrants et de qualité sanitaire des produits.

Actuellement, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation définit l'agroécologie comme une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle s'appuie sur la diversité de nos systèmes de production en vue de préserver notre environnement et nos ressources naturelles. Il s'agit d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production, en maintenant ses capacités de renouvellement. Le présent amendement tend à ce qu'une réflexion soit menée afin de ne pas laisser cette notion majeure sans valeur juridique ou reconnaissance officielle. C'est pourquoi il nous semblerait qu'un décret pourrait utilement élaborer des critères précis à respecter, en termes de croissance de la biodiversité, d'amélioration de la qualité des sols, d'économie d'eau pour l'irrigation, de reconstitution de paysages ruraux de qualité, de réduction des intrants et de qualité sanitaire des produits.

est ainsi libellé : La parole est à M. Henri Cabanel. Il est désormais incontestable que l'agriculture française aura à souffrir prochainement d'un déficit chronique d'alimentation en eau pour l'irrigation, surtout dans les régions méridionales. À ce titre, il faut rappeler que l'alimentation en eau agricole eau agricole pour satisfaire les besoins en irrigation ne peut se faire que de deux manières : par pompage dans les eaux de surface ou par pompage dans les masses d'eau souterraines. Dès lors, une solution privilégiée est de stocker l'eau en période de hautes eaux afin de la restituer en période d'irrigation. Un nouveau procédé, qui constitue une adaptation de la méthode des retenues collinaires, est envisageable : il s'agit de réaliser des stockages d'eau entièrement enterrés, financés par la valorisation des matériaux extraits pour réaliser le stockage, sans faire appel aux finances publiques. L'obligation de recours à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière semble imposer de faire appel aux carriers. Pour éviter de rendre le monde agricole tributaire de la politique commerciale des carriers, une solution a été trouvée une société coopérative d'intérêt collectif- ou SCIC -disposant des capacités techniques nécessaires et totalement indépendante du monde des carriers pourrait être créée. Cette SCIC se chargerait d'obtenir les autorisations d'exploitation. Les travaux de creusement de la réserve et la valorisation des matériaux seraient sous-traités à des entreprises du monde des carriers ou des travaux publics.

territoire et du développement durable ? Cet amendement vise à soustraire les projets d'affouillements du sol nécessaires à la création de réserves d'eau à usage agricole aux prescriptions du schéma régional des carrières. Notre commission avait déjà examiné une telle proposition lors de l'examen du projet de loi pour

De tels affouillements constituent alors techniquement des carrières soumises au régime d'autorisation des ICPE et aux prescriptions du schéma régional des carrières. Malgré la finalité agricole de ces opérations

d'émissions de poussières ou de gestion des déchets. Il en résulterait également une rupture de concurrence avec les carrières, dès lors que les matériaux extraits de ces affouillements pourraient être utilisés à des fins commerciales sans être soumis aux mêmes obligations que les matériaux des carrières. L'avis est donc défavorable. Quel est l'avis

Le présent amendement vise à ce que les surfaces agricoles, dans les aires de protection de captage prioritaires, soient cultivées en agriculture biologique ou selon des modes d'exploitation agroécologiques. Le Grenelle de l'environnement avait identifié, sur le fondement

La feuille de route de la conférence environnementale de 2016 engageait le Gouvernement à renforcer l'effectivité des actions en faveur de leur protection. À ce jour, seulement 43 % de ces captages font l'objet de plans d'action. Le déploiement de l'agroécologie dans ces aires de protection de captage est un objectif prioritaire. Il peut être un levier d'accélération pour le développement des nouvelles pratiques agronomiques.

La protection des zones autour des captages d'eau privilégie une logique partenariale par la mise en place de programmes d'actions élaborés en concertation avec les différentes parties prenantes. Si certains programmes prennent effectivement du temps à mettre en place, c'est souvent parce que la conciliation des différents usages est complexe, comme toujours en matière d'eau. Les études publiées sur ce dispositif soulignent bien qu'il faut privilégier la concertation et la contractualisation. je rappelle que la définition d'une zone soumise à contrainte environnementale reste une option disponible sur décision du préfet pour imposer certaines pratiques agricoles- travail du sol, gestion des intrants, rotation des cultures -lorsque l'approche négociée ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés en temps utile. Ces prescriptions sont toutefois définies en tenant compte des circonstances locales. Imposer dans la loi un pourcentage donné de surfaces consacrées à l'agriculture biologique dans ces zones remettrait en cause cette approche territoriale et négociée. Pour ces raisons,

de l'agriculture à l'eau. Ces ressources doivent pouvoir être mobilisées. Le stockage de l'eau représente une solution durable et pragmatique d'adaptation au changement climatique. Pourtant, malgré de nombreux rapports parlementaires alertant sur la nécessité de développer le stockage de l'eau, les freins existent toujours.

Seule l'alimentation en eau potable de la population bénéficie d'une priorité par rapport aux autres enjeux, ce qui est pleinement justifié par des motifs de santé publique. L'avis est défavorable.

et 168 rectifié visent à accroître la place de l'agriculture au regard des principes de la politique de l'eau. La première partie de ces amendements n'ajoute rien au code de l'environnement, qui prévoit déjà, depuis l'adoption de la loi Montagne du 28 décembre 2016,

: La parole est à M. le ministre. Le développement des énergies renouvelables fait partie des leviers qui permettront de maintenir une agriculture performante en France et d'assurer aux agriculteurs un revenu complémentaire. Cela passe par l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments d'élevage ou le développement de la méthanisation agricole. Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables ne sont possibles qu'à la condition d'être non discriminatoires, transparents et ouverts et de ne pas exclure les entreprises susceptibles de concurrencer des projets en poursuivant le même objectif en matière d'environnement ou d'énergie. Pour ces raisons, le Gouvernement demande la suppression de cet article.

Il s'agit de préciser les modalités du droit à l'injection hors zone de desserte d'un gestionnaire de réseau. Nous souhaitons prévoir dans quelles conditions le raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel des installations de production de biogaz situées sur le territoire d'une commune qui ne dispose pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel est possible. L'amendement n° 569 rectifié ,

nous avons été interpellés sur les conséquences de cette modification apportée par la commission, qui pourrait permettre à un gestionnaire de réseau de distribution de construire des gazoducs pour le raccordement de ces unités de biogaz en dehors de sa zone de concession. Selon ses détracteurs, cette mesure ne prendrait pas en compte le régime des concessions, ne serait pas conforme au droit de la commande publique, pourrait avoir un effet contre-productif en freinant les raccordements en raison d'un risque accru de recours par les communes concernées par ces nouvelles infrastructures et serait susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires en termes de raccordements non justifiés et non optimaux sur le plan économique.

Il n'est bien évidemment pas question de créer un nouveau droit à l'injection absolu. Les limites sont déjà bien définies dans le texte, puisqu'il n'est question que d'installations situées à proximité d'un réseau existant. Elles seront encore explicitées par le biais de deux amendements identiques. En revanche, si le droit ainsi créé devait se limiter aux méthaniseurs méthaniseurs déjà présents dans le périmètre d'une concession, ce qui serait le cas si l'apport de la commission était supprimé, chacun comprend bien qu'on manquerait très largement la cible puisque très peu de méthaniseurs seraient en pratique concernés. Je ne méconnais pas les quelques difficultés juridiques liées au statut des canalisations ainsi créées ; elles sont toutefois très loin d'être insurmontables. Nous avons d'ailleurs travaillé à une rédaction qui a recueilli l'accord du principal gestionnaire de réseaux de distribution, celui de la fédération nationale des collectivités concédantes, la FNCCR, dont chacun connaît la grande vigilance pour défendre les compétences des collectivités en la matière. Cet amendement tend à prévoir que, par dérogation, la canalisation est la propriété du gestionnaire de réseaux, sauf à ce que la commune traversée veuille un jour créer son propre réseau, auquel cas un transfert de propriété serait prévu à sa demande, sur la base d'une compensation encadrée par un décret pris après avis du régulateur. La commission est défavorable aux amendements n 761

de son amendement n° 761 rectifié, qui permet le raccordement à un réseau public de distribution des installations de production de biométhane situées en dehors d'une zone de desserte, tout en préservant la propriété des réseaux publics de distribution de gaz par les collectivités territoriales.

Cet amendement tend à préciser que les conditions et limites qui seront définies par décret visent la pertinence technico-économique des investissements qu'il faudra réaliser pour permettre l'adaptation des réseaux. Il est également nécessaire de prévoir dans les textes la répartition des coûts des adaptations des réseaux entre les gestionnaires de réseaux et les producteurs, ainsi que le principe d'une mutualisation de la part restant à la charge des producteurs entre les différents producteurs qui injecteront dans les réseaux concernés. Il ne faut pas que le premier raccordé supporte l'intégralité de la charge.

notamment les digestats, fabriqués à partir de déchets, hors boues d'épuration. Cela conduit à transformer les méthaniseurs en « machines à laver », notamment des biodéchets, tout en affranchissant les matières en affranchissant les matières produites des obligations auxquelles sont normalement soumises les substances issues de la méthanisation agricole. Cette sortie du statut de déchets qui renvoie toute la responsabilité sur l'utilisateur du digestat, à savoir l'agriculteur, alors que ce dernier rend un service à la société en participant à la gestion des déchets, n'est pas acceptable. Il importe, au contraire, de renforcer l'acceptabilité sociale des méthaniseurs, de préserver l'environnement et les sols au moment de l'épandage des digestats et de participer à la montée en gamme de l'agriculture française. Aussi, pour sécuriser la filière méthanisation, est-il essentiel de revenir sur cet ajout en supprimant l'article 16 D. Quel est l'avis de

: les matières concernées devront être conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté, un règlement européen ou un cahier des charges approuvé par voie réglementaire et remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, dont l'absence d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. Concrètement, et même s'il était déjà possible d'épandre des digestats sur les sols agricoles, cette sortie du statut de déchets vise à améliorer l'image de l'épandage des digestats et, indirectement,

Comme cela a été rappelé en commission, il est déjà possible d'alimenter les méthaniseurs par toute une série de matières, qu'elles proviennent de traitements des eaux usées, de stations d'épuration, d'activités agricoles ou d'industries agroalimentaires, selon des règles

tel que prévu par l'article 16 D, et, d'autre part, à s'assurer que la valorisation au sol de matières fertilisantes ou supports de culture reste soumise au respect d'un plan d'épandage visé par l'autorité administrative compétente.

Il apparaît donc nécessaire de compléter la rédaction de cet article pour y faire référence et sécuriser davantage encore le dispositif de sortie du statut de déchets. Enfin, si ce dispositif soumet les matières en question au respect des cahiers des charges existants,

Ce dispositif est conforme aux solutions mises en oeuvre ces dernières années sous l'égide du ministre Stéphane Le Foll, notamment la publication d'un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes. La poursuite des discussions avec le ministre de l'agriculture doit donner lieu à la publication de deux nouveaux cahiers des charges, conformément aux engagements pris.

l'utilité du CORENA est reconnue. Cette instance permet d'assurer le partage en amont de l'information et des impacts technico-économiques des réglementations, d'éviter les incohérences ou les redondances entre les réglementations et d'en faciliter la mise en oeuvre ultérieure par les agriculteurs et les services de l'État.

Sa mission est essentielle aujourd'hui pour simplifier les normes pesant sur nos exploitations et éviter toute surtransposition. L'article précise ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement. C'est une consécration législative pour ce comité reconnu par la profession et que le Parlement pourra dès lors contrôler.

la protection des filières de race française, garantie de qualité et de traçabilité des produits offerts à la consommation, en lien direct avec le titre II de ce projet de loi. En effet, cette traçabilité, inhérente au savoir-faire et à la tradition de nos filières de viandes, est synonyme d'une alimentation saine et de qualité pour les consommateurs. Le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution précise que tout amendement est recevable dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Pour ce qui concerne mon amendement, le lien direct existait. Les services de la commission ont bien tenté d'augmenter l'irrecevabilité à partir d'une partie de l'amendement qui se contentait de reprendre mot pour mot le code rural et de la pêche maritime tel qu'il est écrit. Les modifications concernaient les articles situés avant et après le passage évoqué.

les services de la commission ont fini par nous conseiller de détourner la procédure parlementaire, en prenant la parole sur n'importe quel article pour obtenir une réponse du ministre. On se retrouve dans une situation où, pour remédier à leur propre désinvolture, nos services, madame la présidente de la commission, nous conseillent de détourner la procédure parlementaire et d'aller à l'encontre des usages admis dans cette assemblée ! Ce cas de figure s'est déjà produit un peu plus tôt pour un autre amendement déposé par les sénateurs de la République En Marche, l'amendement

le monde agricole voulait bien faire crédit, quelque temps, au regard des bonnes intentions affichées et des objectifs que chacun ne pouvait que partager : redonner du revenu aux producteurs et améliorer la qualité alimentaire, sans jamais préciser qui allait devoir payer. Après des dizaines d'heures de travail dans des conditions regrettables faute de pouvoir y consacrer le temps voulu, notamment en commission, deux sentiments se sont installés : le scepticisme et la déception. Scepticisme quant à ce que produira effectivement la nouvelle économie mixte que vous avez inventée, ce mélange d'économie administrée à coup d'indicateurs, dont nous sommes bien curieux de voir à quoi ils aboutiront pour les producteurs en manque de poids économique, et de libre marché, qui permettra toujours aux grands acheteurs d'aller voir ailleurs si les prix ne leur conviennent pas ou si leurs marges se dégradent. À moins que les consommateurs français ne paient le regain de valeur ! Nous serions alors dans un non-dit de grande portée politique, que nous ne saurions approuver. En définitive, avec ce titre I, il s'agit d'aménagements de lois votées précédemment ; rien de plus, rien de moins ! À cela s'ajoute notre profonde inquiétude que les hypothétiques bénéfices de cette loi soient annihilés par la baisse annoncée du budget de la PAC. Sur ce sujet, nos inquiétudes restent vives. Pour ce qui est du titre II, les déceptions sont grandes par rapport à la nécessité de la prise en compte des fortes attentes de la société. Pour un peu, les 20 % de bio dans la restauration collective disparaissaient ... Que dire de la suppression des dispositifs visant à interdire l'utilisation du terme de gratuité comme outil promotionnel, à introduire des exigences environnementales dans les cahiers des charges des SIQO, alors même que le délai envisagé est de 2030, à encadrer davantage l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ? Que dire du refus du Gouvernement et de la majorité sénatoriale de reconnaître dans la loi l'importance de l'agriculture de groupe ? Que dire de leur opposition systématique aux amendements ayant pour objet l'agroécologie, ou encore de leur refus d'interdire la déforestation importée ? ? Finalement, que penser du rejet de la quasi-totalité de nos amendements visant à renforcer la qualité alimentaire des repas servis dans la restauration scolaire ou collective, à interdire la publicité pour les aliments transformés à destination du jeune public, à à mettre en place des objectifs clairs en matière de réduction du sucre, du sel et du taux de matière grasse dans les aliments et à renforcer l'étiquetage des denrées alimentaires ? Ainsi, seulement 10 amendements de notre groupe sur les 140 que nous La coconstruction n'a pas eu lieu ! Une satisfaction, néanmoins : l'adoption du Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytosanitaires. Tout de même ! Pour conclure, le bilan de ce texte est pour notre groupe très décevant, très en deçà du minimum que les agriculteurs et les Français, en tant que consommateurs, étaient en droit d'attendre de nous. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre

Les États généraux de l'alimentation avaient abouti à une rédaction permettant à tous les maillons de la chaîne alimentaire de prendre leurs responsabilités. Or, après son examen par notre chambre, le texte est dénaturé. Sa première partie ne correspond plus à la philosophie initiale des États généraux de l'alimentation. Tandis que nous souhaitions que les interprofessions se coordonnent, s'organisent et se responsabilisent pour un partage de la valeur plus juste,

Tandis que nous souhaitions refonder, après concertation, le statut des coopératives pour plus de transparence entre les associés coopérateurs et leur structure, la majorité sénatoriale a fait le choix du. Tandis que Tandis que nous proposions une refonte environnementale de notre modèle agricole, l'une des mesures clés du projet présidentiel, à savoir la séparation capitalistique du conseil et de la vente des produits phytosanitaires, La seconde volonté des auteurs de ce projet de loi était de répondre aux attentes sociétales, au travers d'une alimentation saine et durable. Mes chers collègues, au cours de nos débats, nous avons su trouver des positions de compromis, afin d'améliorer le texte. Je pense, par exemple, à la mise en place du formalisme lors des négociations commerciales entre distributeurs et industriels, à la faculté des parlementaires de saisir l'ANSES, ou encore à l'élargissement de l'expérimentation de la pulvérisation par drones. Nous nous félicitons également de la sagesse du Sénat, qui, en séance publique, a finalement adopté deux mesures clés du projet de loi : le rétablissement de l'objectif de 20 % de produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective et l'élargissement du champ d'application de l'interdiction des néonicotinoïdes. Ce sont des avancées non négligeables, permettant de conserver l'esprit des États généraux de l'alimentation et répondant à une attente sociétale forte. Enfin, mes chers collègues, j'aimerais me féliciter des débats et des échanges que nous avons eus. Les sujets que nous avons abordés ces derniers jours étaient importants pour l'avenir de nos filières, pour le quotidien de nos agriculteurs et pour l'alimentation des Français.

Nous partageons les objectifs des auteurs du projet de loi. Comment, en effet, ne pas souscrire à l'impérieuse nécessité de rééquilibrer les relations commerciales agricoles ? À cet égard, les améliorations apportées par la Haute Assemblée méritent d'être soulignées ; je pense notamment à l'encadrement du choix des indicateurs, au renforcement du médiateur des relations commerciales agricoles ou encore à la précision de la revente à perte et aux limitations des offres promotionnelles. Toutefois, comme nous l'avons souligné, cela ne sera pas suffisant pour moraliser les négociations commerciales. Mes chers collègues, comment ne pas défendre une exigence minimum de qualité et de sécurité des produits dans la restauration collective publique ? Même si nous pouvons nous satisfaire de la réintroduction de l'objectif de 20 % de produits bio dans la restauration, bio dans la restauration, nous ne pouvons que regretter la faiblesse des sanctions en matière de rappel et de retrait de produits, alors que nous sortons à peine du scandale Lactalis Enfin, comment ne pas défendre l'idée qu'il faut réduire drastiquement l'utilisation de pesticides sur notre territoire ? Si nous nous réjouissons de la reconnaissance d'un fonds d'indemnisation des victimes professionnelles des produits phytopharmaceutiques, nous ne comprenons pas la frilosité de la majorité du Sénat sur la remise en cause des rabais et ristournes en matière de PPP ou sur l'interdiction du glyphosate.

Si nous voulons sauver l'agriculture française, l'amener vers plus de qualitatif, il faut des prix minimaux garantis. Il est insupportable de se cacher derrière le droit à la concurrence européen tout en le dénonçant ! Or cela fait trente ans que l'agriculture est la variable d'ajustement de la guerre des prix, au nom de la concurrence libre et non faussée. Vous l'aurez compris, notre groupe ne votera pas ce texte.

des relations plus équilibrées au profit des agriculteurs. Je pense à l'inversion de la construction des prix, à la contractualisation, à l'aide d'indicateurs de coûts de production,

les points majeurs figure effectivement la relocalisation de l'approvisionnement de la restauration collective. Notre groupe se satisfait de la réintégration des 20 % de produits

pour l'avenir du secteur agricole, dans sa diversité. Les modalités adoptées sur la construction du prix pour redonner aux producteurs leur place

Le scrutin est ouvert.

cohérente avec la politique agricole commune ! Oui, nous devons avoir une politique de concurrence permettant que nos produits ne subissent pas de concurrence déloyale au sein de nos frontières européennes ! C'est un travail de longue haleine, mais nous le menons mais nous le menons avec toute la volonté et toute la détermination que vous pouvez nous connaître. Il reste à construire des trajectoires pour tirer notre agriculture vers le haut, vers l'innovation, vers plus d'audace, vers la simplification et vers cette montée en gamme que nous appelons de nos voeux. Le texte essaye de répondre à cette problématique. Ce n'est pas une loi d'orientation agricole. Cela fait partie de la politique de l'alimentation que nous souhaitons mettre en place entre 2018 et 2019. C'est une brique, et nous contribuons ainsi à construire le mur de cette agriculture, avec des fondations solides.